D'abord, les sous-secteurs mentionnés dans le texte ne sont pas définis. Or l'information donnée serait de nature très différente selon les sous-ensembles retenus. Ensuite, cet affichage serait en réalité peu cohérent avec le champ des lois de financement de la sécurité sociale, qui ne comprend pas ces régimes. Par ailleurs, cette présentation serait compliquée par le fait qu'une partie des dépenses du champ des ASSO, notamment les régimes obligatoires de sécurité sociale, est suivie en comptabilité générale et non en comptabilité nationale. Enfin,

texte. Quel est l'avis de la commission ? Le fait même que le rapport économique, social et financier fournisse une telle information montre bien que l'administration est tout à fait capable de la produire. De plus, il serait utile de disposer de ce degré de précision- je le dis pour mes collègues -, si, à l'avenir, il fallait expliquer les écarts entre les prévisions

à l'assurance chômage. Cette mesure, adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat, figurait dans le texte initial du député Thomas Mesnier, qui voulait intégrer les comptes du régime de l'assurance chômage dans le projet de loi de financement de la Si cette disposition ne figurait plus dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, c'est en raison de l'opposition de l'ensemble des organisations syndicales et patronales. La proposition d'inclure ce régime dans le champ du PLFSS remet en cause sa gestion paritaire. sa gestion paritaire. Le député Mesnier l'a appris à ses dépens puisqu'il a dû retirer l'assurance chômage du texte à la suite de l'accomplissement d'un miracle : la rédaction d'une déclaration d'opposition commune du Medef et de l'ensemble des syndicats En intégrant l'assurance chômage dans la loi de financement de la sécurité sociale, la loi organique modifierait irrémédiablement la gouvernance et la nature de ce régime. Elle rendrait sa gouvernance encore plus complexe en réduisant de nouveau la place des partenaires sociaux. La gestion La gestion du régime par les organisations syndicales et patronales est un pilier de la démocratie sociale, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, et ne saurait être remise en cause

n° 13 rectifié. La commission des affaires sociales du Sénat, sur proposition du rapporteur, veut étendre le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale à l'assurance chômage.

Par ailleurs, pendant la crise de la covid, l'Unédic a joué son rôle d'amortisseur social. Or la crise sanitaire, avec ses conséquences sociales, est malheureusement loin d'être terminée. Réduire les prérogatives des partenaires sociaux ne nous paraît donc ni justifié ni pertinent.

Il vise à supprimer l'extension du champ des lois de financement de la sécurité sociale à l'assurance chômage et à rétablir la version du texte adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Les différents intervenants l'ont souligné, le régime d'assurance chômage fait l'objet d'une gestion paritaire particulière. On peut comprendre

Cet amendement vise à supprimer, d'une part, la possibilité de fixer des crédits limitatifs, et, d'autre part, l'instauration de ratios obligeant à une ratification des crédits supplémentaires qui seraient ouverts par décret en cas de dépassement. Cette double suppression nous paraît nécessaire afin de préserver la nature de l'Ondam,

sociale fixent [ ...] ses objectifs de dépenses ». La loi organique ne peut donc prévoir l'introduction de crédits limitatifs dans l'Ondam et doit laisser à la loi ordinaire le soin de prévoir des mécanismes d'encadrement de la dépense. Par ailleurs, l'introduction de ratios au-delà desquels une procédure de ratification est enclenchée vise, certes, à encadrer les dépenses d'Ondam, mais elle est redondante avec le rôle du comité d'alerte. Il est déjà prévu que, en cas de risque de dépassement de l'objectif supérieur à 0,5 %, le comité doit prévenir le Parlement Cette procédure d'alerte indépendante est la plus adaptée, nous semble-t-il, au fonctionnement des dépenses de santé. De plus, il est contraire au caractère transversal de l'Ondam de déclencher une telle procédure en cas de dépassement du ratio sur un seul des sous-objectifs. tel mécanisme entraînerait en réalité une rigidité excessive au sein même de l'Ondam, dont le pilotage serait désormais différencié entre ses différentes composantes, sans pour autant offrir les outils de maîtrise des dépenses adaptés. Concrètement, le texte, tel qu'il résulte des travaux de la commission, risquerait de nourrir un antagonisme entre médecine de ville et médecine hospitalière, alors que les deux sont complémentaires. L'encadrement plus strict que vous proposez, s'agissant du sous-objectif de l'Ondam hospitalier, ne manquerait pas d'être perçu comme une forme de suspicion à l'égard de l'hôpital. d'autant plus malvenu, me semble-t-il, et je sais que vous en êtes d'accord, au sortir d'une crise sanitaire qui a vu l'hôpital être en première ligne. Par ailleurs, nous vous proposons de modifier le texte sur la non-contraction des recettes et des dépenses. Le texte issu des travaux de la commission supprime la possibilité de telles contractions, en mettant notamment en avant la contribution des organismes complémentaires qui a été votée l'an dernier. Il était pourtant parfaitement logique que cette contribution vienne atténuer l'Ondam, dans la mesure où il s'agissait de dépenses pour lesquelles la sécurité sociale s'était substituée aux complémentaires, qui, en temps normal,

à la sécurité sociale sur les prix de produits pharmaceutiques. Interdire de les prendre en compte reviendrait à afficher une dynamique de l'Ondam plus importante que la réalité, décorrélée de l'évolution effective des dépenses, et qui s'éloignerait de son rôle de pilotage des dépenses de santé et

Mme Raymonde Poncet Monge. Depuis l'instauration de l'Ondam, la dotation accordée aux hôpitaux publics par les gouvernements successifs a systématiquement été inférieure à l'évolution des besoins de santé et, conséquemment, au coût des soins hospitaliers.

cette logique financière étrangle l'hôpital et concourt à la dégradation des soins et des conditions de travail des soignants. L'endettement des structures hospitalières qui en découle entrave les investissements nécessaires à l'exercice de leur mission de service public. Or, s'il apparaît nécessaire d'utiliser un outil et des indicateurs de suivi des dépenses, ce n'est pas la logique comptable de court terme qui doit dicter le niveau des dépenses de santé. C'est, bien davantage, une décision démocratique

visant à établir les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, afin de leur donner plus de visibilité. La loi de financement de la sécurité sociale de 2020 a prévu qu'un protocole entre l'État et les fédérations représentatives des établissements de santé publics et privés puisse établir les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles de ces établissements et les engagements réciproques afférents. Le premier protocole a été conclu pour la période allant de 2020 Dans son dernier rapport, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie estime néanmoins que les éléments actuels de pluriannualité sont insuffisants et qu'ils souffrent d'un manque de visibilité et de cohérence. Il recommande l'élaboration d'une trajectoire à cinq ans des objectifs,

même si, on est bien d'accord, celui-ci aurait tout intérêt à se renouveler. Je l'ai dit hier, nous sommes à la disposition des partenaires sociaux pour réfléchir, avec eux,

et qui, à mon avis, se méprend sur les intentions du constituant de 1996. Le garde des sceaux de l'époque, Jacques Toubon,

Sans remettre en cause l'approche particulière des assurances sociales, nous voulons tirer les conséquences, comme Corinne Imbert l'a d'ailleurs rappelé lors de la discussion générale, de ce qu'est l'Ondam aujourd'hui, à savoir un mélange de dépenses relevant d'assurances sociales et de dépenses d'intervention. Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution prévoit bien que les objectifs de dépenses sont votés « dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique organique ». Le Conseil d'État, certes réservé sur le concept de crédits limitatifs, a souligné que l'absence de caractère limitatif des crédits ne faisait pas obstacle à ce que le législateur organique puisse définir les modalités d'information ou de saisine du Parlement en cours d'exécution d'une loi de financement de la sécurité sociale. C'est donc bien de ces modalités, et des conditions et réserves mentionnées à l'article 34 de la Constitution, que relève le dispositif

et que vous ne considérez pas comme contraires à l'article 34 de la Constitution. Ne travestissons pas les modifications que nous entendons porter à la construction de l'Ondam

Ne prétendez pas non plus que les hôpitaux se verraient dans l'incapacité d'accueillir des patients ou que les achats de masques en urgence auraient été rendus impossibles en 2020, du seul fait que nous aurions demandé l'avis de la commission Au contraire, permettez-nous de considérer que les dépenses de santé sont stratégiques et qu'il est du devoir du Parlement de vouloir en débattre et, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous le prescrit, d'en « constater la nécessité » et d'en

L'intention de ses auteurs est de dénoncer le sous-financement du système de santé, mais cette rédaction ne me paraît ni opérationnelle ni pertinente. Par définition, l'Ondam que nous votons s'appuie sur le tableau sanitaire et social que nous dressons de notre pays et sur les besoins que nous identifions. La commission émet donc un avis défavorable

nous l'appliquons. Je rappelle que, au-delà des financements complémentaires apportés par le Ségur de la santé- 12,5 milliards d'euros en 2022 -, la progression de l'Ondam hospitalier en base sera de 2,7

Madame Cohen, d'assurance maladie est pour le moins paradoxal ... Chaque année, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les parlementaires que nous sommes

ni des ratios obligeant à une ratification des crédits supplémentaires au-delà d'un certain seuil, mais seulement des objectifs ». De deux choses l'une : soit l'Ondam est un simple objectif et, par conséquent, les parlementaires comme les établissements de santé peuvent augmenter les dépenses au-delà de cet objectif, si les besoins le justifient ; soit l'Ondam est un plafond indépassable et le Gouvernement doit rendre des comptes devant le Parlement lorsque les dépenses sont supérieures à celles qui

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a précisé que le monopole des lois de financement de la sécurité sociale sur les mesures d'exonération concernerait uniquement les exonérations non compensées par l'État.

Mais, au-delà du principe, ce qui nous pose problème, ce sont les montants concernés. Pour rappel, de 2011 à 2017, les exonérations de cotisations patronales

derrière le mot « transparence », se cache l'organisation de l'assèchement des recettes de la sécurité sociale. Les choix budgétaires arrêtés conduisent à l'austérité de notre système de protection sociale et à la dégradation de nos services publics. Quel

l'intention initiale de notre collègue député Thomas Mesnier : interdire l'adoption de toute mesure de réduction de ressources de la sécurité sociale d'une durée de plus de trois ans, même compensée, en dehors d'une loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agissait là d'un principe simple,

Ces cadeaux faits aux entreprises sont autant de recettes en moins pour la sécurité sociale ; j'y insiste, nous parlons de milliards d'euros ! Or nous sommes assez nombreux dans cet hémicycle à dénoncer la non-compensation de ces exonérations par l'État depuis 2018.

Bien sûr, les dépenses ont augmenté avec la crise sanitaire ; mais, dans ce cas, mettons fin aux exonérations pour éviter de creuser le déficit. Les non-compensations se sont multipliées, pour un coût réel de plus de 4 milliards d'euros par an, et ce uniquement depuis 2018, année où le gouvernement d'Édouard Philippe a choisi de remettre en cause ce principe fondateur. On a donc beau jeu, trois ans après, de prétendre refonder le financement de la sécurité sociale sans lui donner les moyens d'assurer ses missions et de répondre aux besoins.

; en parallèle, 1,6 milliard d'euros seront consacrés à l'enseignement scolaire en 2022. Pour reprendre le titre du livre de mon ami Éric Bocquet, on parle bien là de « milliards en fuite ».

Cela étant, nous ne nous contentons pas de dénoncer : nous proposons, par cet amendement, de créer un principe de non-prolifération des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Tout nouveau dispositif entraînera la suppression d'un dispositif existant pour un montant équivalent.

Même avis.

entre l'encadrement des exonérations et la liberté du législateur ordinaire, à laquelle je ne doute pas que vous êtes très attachée. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

disposition est inconstitutionnelle. Or, en vertu de la Constitution, « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues

dire ! Quel est l'avis de la commission sur les amendements n

Actuellement, ce contrôle est limité par le secret des affaires. Or, dans le contexte actuel d'inflation du prix des médicaments et de pandémie de covid-19, il est plus que jamais essentiel de progresser en faveur de la transparence des prix des médicaments. À cet égard, je rappelle l'engagement des parlementaires communistes lors de la campagne européenne pour la levée des brevets

dire ! Quel est l'avis de la commission sur les amendements n

l'amendement n° 1 rectifié. Cet amendement vise à compléter le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale par un prévisionnel consacré aux médicaments,

des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir cette disposition n'introduit pas de véritables contraintes dans la rédaction de ce rapport. Lors des travaux préparatoires de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, à l'origine des dispositions imposant un rapport pluriannuel, il a été relevé qu'« aucune limite autre que celle de l'objectif d'équilibre à moyen terme des comptes de l'ensemble des régimes n'est posée à la détermination par le Parlement des orientations à moyen terme des dépenses et des recettes de la sécurité sociale

« en termes de contenu, le nouveau rapport exigé se limite plus rigoureusement que le précédent rapport aux seules questions de financement de la sécurité sociale ». La pluriannualité que ce rapport est censé instituer reste donc on ne peut plus limitée. Cette vision à court terme des dépenses de santé semble bien décalée, au moment même où la crise sanitaire nous impose de rendre aux acteurs du système de santé une certaine visibilité.

Le défaut de visibilité et l'instabilité juridique subséquente constituent des facteurs reconnus de la perte d'attractivité de la France auprès des investisseurs industriels. Aussi, cet amendement tend à enrichir le rapport existant en y introduisant une dimension pluriannuelle relative au budget du médicament,

a inséré un indicateur supplémentaire : la mesure du solde entre les dépenses et les recettes de la sécurité sociale. Derrière cet outil se cache la volonté de mettre en exergue les dépenses jugées excessives de la sécurité sociale par rapport aux recettes, amputées chaque année de près de 100 milliards d'euros d'exonérations et de réductions de cotisations. Surtout, avec la création de cet indicateur, de transposer les règles des soldes structurels de la Commission européenne, lesquelles imposent aux États européens de ne pas dépasser un déficit de 3 % et un taux d'endettement de 60 %. Cette volonté est assumée par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin. l'a confirmé lui-même : l'objectif est « de faire du printemps, à l'occasion de la transmission du programme de stabilité à la Commission européenne, le grand moment parlementaire de débat d'orientation des finances publiques ». Nous refusons cette logique d'austérité dictée par l'Europe et, en conséquence, nous demandons la suppression du solde dans les indicateurs de la sécurité sociale. L'amendement L'article 2 ajoute aux lois d'approbation des comptes de la sécurité sociale une annexe présentant une évaluation des politiques de sécurité sociale relatives à chaque branche, rappelant les objectifs assignés, les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre. Or cette disposition est problématique, singulièrement pour ce qui concerne la branche vieillesse et l'annexe chargée d'analyser l'évolution de la soutenabilité financière de l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires

ce mécanisme d'équilibre pluriannuel automatique entre les dépenses et les recettes est en réalité une généralisation de l'Ondam aux comptes de la sécurité sociale.

même logique qui a conduit à fermer des hôpitaux, à supprimer 100 000 lits en vingt ans, à annuler les projets d'investissement, à imposer un insuffisant pour répondre aux besoins et, globalement, à dégrader les conditions de travail et de rémunération des personnels hospitaliers, ainsi une pénurie de personnels. En réalité, cette règle d'or est un arrêt de mort pour les hôpitaux. Nous refusons cette obsession de réduction des dépenses sociales,

tout en préservant évidemment les capacités d'action de la sécurité sociale comme stabilisateur économique. Par conséquent, s'imposer de présenter des comptes sociaux à l'équilibre dès 2025, comme vous le proposez- qui plus est sans indiquer les moyens permettant d'y parvenir -nous condamnerait soit à prévoir de façon précipitée des mesures allant à l'encontre la politique menée par le Gouvernement soit à nous fixer un objectif peu crédible. Nous excluons donc de procéder à des coupes claires, aveugles, notamment dans notre système de santé, en faveur duquel nous avons consenti des efforts inédits depuis 2017 et dont la crise a révélé toute l'importance. De même, alors que la croissance redémarre, il serait irresponsable de risquer de la briser dès maintenant par une réduction drastique de l'investissement et du soutien publics. Vous vous en souvenez, le précédent de la crise de 2008 a montré combien il était contre-productif d'engager une politique de redressement des comptes trop brutale. C'est la croissance

sécurité sociale. Ces PEPSS ont pour but, selon le rapporteur, d'offrir une meilleure vision de la structure des dépenses à venir de chaque branche

Tout d'abord, ces indicateurs, comme les soldes budgétaires, mesurent uniquement les recettes et les dépenses, sans prendre en compte l'ensemble des conséquences positives des dépenses sociales. À titre d'exemple, la hausse des salaires des personnels de l'aide à domicile

bien les limites de ces mécanismes budgétaires borgnes et déshumanisés. Enfin, ces programmes d'efficience font la part belle à celles et ceux qui veulent segmenter les branches de la sécurité sociale et les rendre toujours plus étanches, alors que la sécurité sociale est une maison commune. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces PEPSS.

de la sécurité sociale nouvellement créé détaille les annexes qui seront jointes au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, notamment celles qui présentent les rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche. Il précise que ces rapports s'appuient sur « un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l'exposé des résultats atteints lors des dernières années Cet amendement vise à préciser que cet exposé concernera les résultats atteints lors des trois dernières années, afin de garantir la qualité et la pertinence des analyses qui en seront tirées.

L'article 2 prévoit que les rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale annexés au projet de loi d'approbation comprennent désormais une analyse de « l'évolution de la soutenabilité financière

La commission a, au contraire, souhaité que les éventuels écarts par rapport aux prévisions de la loi de programmation

des finances publiques, d'autre part, la création d'une annexe informative sur les régimes complémentaires. Contrairement à ce que craignent les auteurs de cet amendement, une telle amélioration de l'information du Parlement ne remet en aucune façon en cause la gestion paritaire. Nous nous

la description de ses intentions est de nature à éclairer le Parlement. Il convient donc de conserver ce dispositif, en rejetant cet amendement. Je rappelle d'ailleurs que la commission a complété le compteur des écarts introduit par les députés. Les écarts, et donc les mesures, concerneront aussi les recettes-

L'instauration d'un mécanisme permettant de couper le robinet de la dette sociale sera nécessaire lorsque la crise actuelle sera derrière nous. À cet d'État, je redis ma disponibilité pour discuter des modalités précises de la règle d'or ou encore de sa date d'entrée en vigueur. En effet, vous avez l'air de dire que 2025, c'est un peu tôt.

Je regrette que cet amendement vise à affaiblir cette information sous prétexte que la commission voudrait réduire les dépenses sociales. Nous voulons simplement en mesurer l'intérêt et l'efficience,

vertueux que le Gouvernement entend reprendre en loi de finances par la création des lois d'approbation dissociées des LFSS. J'entends que cela surchargerait l'administration.

Concrètement, pour prendre l'exemple des retraites, il serait bon, comme cela est fait pour le bleu budgétaire du compte d'affectation spéciale « pensions », de savoir combien de nouveaux retraités sont attendus pour l'année à venir, quel serait le niveau de la pension moyenne et comment s'explique l'évolution de la dépense.

le Gouvernement se soit senti obligé de remonter à la création des lois de financement de la sécurité sociale, mais cette précision rédactionnelle n'est pas nuisible ! Sans enthousiasme, bien sûr, la commission émet un avis favorable

analyse l'évolution de la soutenabilité financière de l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévisions et les déterminants de l'évolution à long terme des dépenses, des recettes et des soldes de ces régimes. Il me semble que la présentation d'une telle analyse contribuerait à éclairer le Parlement sur la situation financière globale du système des retraites, sans pour autant remettre en cause la gestion autonome des régimes complémentaires

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier »- non de son déséquilibre permanent ! - « et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses. » C'est ce qui C'est ce qui est dit dans la Constitution, madame Apourceau-Poly ! On peut vouloir changer les termes de la Constitution, mais je ne pense pas que tel soit l'objectif d'une loi organique. Enfin, tout ceci s'inscrit dans des lois de programmation pluriannuelle, ces orientations pluriannuelles s'inscrivant « dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques

conséquent, vous allez continuer d'affaiblir notre système de sécurité sociale et l'orienter encore davantage vers un financement par l'impôt.

d'augmenter les recettes. Je dis simplement qu'il est de notre devoir de respecter l'équilibre pour les générations futures. Voilà ce qu'est la règle d'or. Je

Le scrutin est ouvert.

Lorsque des évaluations aboutissent à constater l'inefficacité de certaines niches, celles-ci ne sont que fort rarement remises en cause. Or il ne s'agit pas de quelques euros, mais de milliards d'euros. Il est donc indispensable que la représentation nationale puisse avoir une connaissance plus fine de l'utilisation par les entreprises de ces dispositifs. Pour favoriser la transparence, nous proposons de disposer d'une évaluation précise et détaillée de l'impact des mesures d'exonération sur les créations d'emplois et les dynamiques salariales au sein de cette annexe. Puisque vous êtes favorables aux exonérations, voyons au moins si elles sont efficaces

un coût moyen de 180 000 euros par emploi. Dans la mesure où le coût moyen pour un emploi en France est de 40 000 euros, mes chers collègues, vous jugerez de l'efficacité

Quel est l'avis de la commission sur les amendements

Cette revendication de justice sociale par les organisations syndicales, dont la CGT, est donc efficiente en matière d'équilibre des comptes sociaux.

nous savons imparfait, car il est déconnecté de l'évolution tendancielle des besoins de santé de la population. L'enveloppe financière destinée aux hôpitaux reste la principale variable d'ajustement sur laquelle les gouvernements successifs pour comprimer les dépenses de santé, faute de pouvoir maîtriser les dépenses de médecine de ville. Le résultat en est une réduction de l'offre publique hospitalière sur le territoire Pour notre part, nous estimons que la construction de l'Ondam doit davantage prendre en compte les besoins de santé de la population et l'exigence d'égalité d'accès aux soins dans les territoires. Dans cette logique, le présent amendement vise à intégrer au sein de l'annexe relative au périmètre de l'Ondam une analyse de son évolution au regard du principe d'égalité d'accès aux soins. Quel

Mme Raymonde Poncet Monge. Dans un contexte d'inflation du prix des médicaments qui menace la soutenabilité de notre système de santé,

il est essentiel de progresser sur la question de la transparence du marché pharmaceutique, en vue de renforcer notre démocratie sanitaire et de garantir l'accès aux produits de santé pour toutes et tous. lors, il convient de créer un document budgétaire retraçant les dépenses effectuées par l'assurance maladie dans ce domaine, qui permette aux parlementaires d'avoir accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de leur fonction de contrôle des dépenses sociales. En effet, les PLFSS- en particulier leur annexe 7

ne permet pas de reconstituer le montant détaillé et exhaustif des économies imputables aux médicaments, qui sont disséminées dans les différents sous-objectifs de l'Ondam. L'ajout aux LFSS d'une nouvelle annexe consacrée aux médicaments permettrait de retracer en toute transparence le budget que la France alloue aux médicaments.

Dominique Théophile. Cet amendement vise à supprimer l'obligation d'annexer aux PLFSS le détail de la structure de financement des établissements de santé et, pour chaque région et chaque établissement, le détail et les finalités de chaque dotation reçue.

permanence de soins, recherche, etc. et mieux appréhender les dépenses d'investissement. Dans la mesure où cet amendement tend à revenir sur la position de la commission, celle-ci émet un avis défavorable.

qui en évalue l'impact financier et l'efficacité au regard des objectifs visés. Cet apport constitue une avancée vers plus de transparence. Le recours aux exonérations de cotisations dans le cadre des politiques de baisse des prélèvements obligatoires est devenu courant et croissant, alors que le Parlement n'est qu'insuffisamment informé sur leur véritable impact et leur efficience, en particulier sur la compétitivité des entreprises ou sur le marché de l'emploi. De plus, ces exonérations ne sont pas sans effet sur les comptes des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement. D'un côté, certaines mesures,

Cet amendement vise à préciser que les délais constitutionnels encadrant l'examen des PLFSS par le Parlement ne s'appliquent qu'au PLFSS de l'année, à l'exclusion des projets de loi de finances rectificative et des projets de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Quel

L'Assemblée nationale a introduit une disposition aux termes de laquelle la conférence des présidents de chaque assemblée pourra décider de consacrer prioritairement une semaine au contrôle de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale. Il s'agit d'élever au rang organique le Printemps de l'évaluation qu'organise chaque année l'Assemblée nationale, à l'instar de l'article 8 de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. le Conseil d'État considère que cette disposition établit une procédure pour laquelle la Constitution ne prévoit pas de renvoi à une loi organique ; il recommande donc sa suppression. La commission des finances l'a ainsi supprimée lors de l'examen de la proposition de loi relative à

depuis la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les deux assemblées ont chacune créé en leur sein une mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale afin de suivre et de contrôler l'application des LFSS et de procéder à l'évaluation de toute question touchant aux finances de la sécurité sociale. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer l'inscription du Printemps de l'évaluation dans la loi organique.

de l'arrêt du Conseil d'État, monsieur Fialaire. En effet, si la Constitution ne prévoit pas de loi organique pour une telle procédure, elle ne dit pas qu'il soit inconstitutionnel d'en prévoir une. Il nous semblait intéressant de pérenniser un dispositif objectif et constructif d'évaluation

de la Constitution en ce qui concerne le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale et la certification de la régularité et de la fidélité des comptes du régime général.

la réalisation des enquêtes demandées par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que la production du rapport sur l'application des LFSS et du rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale.

Mme Florence Lassarade. Une loi de programmation pluriannuelle de la santé permettrait de réinjecter une dimension plus prospective dans le débat sur les dépenses de santé, tout en prévoyant des orientations budgétaires à plus long terme.

laquelle dresserait les grandes orientations de la France en matière de santé et les moyens financiers déployés en parallèle pour y répondre.

le champ des PLFSS. Ces modifications n'ont malheureusement pas été adoptées par notre assemblée et nous le regrettons. Nous espérons que le travail de consensus empreint de responsabilité qui animera la commission mixte paritaire permettra de revenir sur certaines dispositions. Nous partageons tous le souhait de voir les lois de financement de la sécurité sociale renforcées ; il serait dommage de créer un cadre si contraignant qu'il limite leur portée. Pour autant, parce que les textes qui nous sont présentés sont rares et importants,

Le scrutin est ouvert.

parole est à M. le secrétaire d'État. Par cet amendement, le Gouvernement propose de revenir sur la modification de la procédure d'avis rendu par les caisses de sécurité sociale, qui a été introduite en commission. Pour rappel, la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale permet une refonte substantielle de la procédure actuelle : les avis seraient désormais remis directement au Parlement et non plus au Gouvernement, et les caisses disposeraient désormais d'un délai plus long pour rendre leur avis. Or la commission propose que les avis soient rendus sur l'avant-projet de loi et non sur le projet de loi lui-même, ce qui ne nous apparaît pas souhaitable pour au moins trois raisons que je vais exposer. Tout d'abord, dans la mesure où l'avis serait rendu après le dépôt du projet de loi, il n'est pas utile qu'il soit remis sur l'avant-projet de loi : cet avant-projet serait de fait, et par construction, déjà caduc.

L'essentiel est en effet que l'avant-projet de loi soit transmis en même temps que le projet de loi. Ce qui nous importe est que nous puissions avoir l'information en direct, le plus rapidement possible.

le constat qui m'amène ici est simple et je ne doute pas que vous le partagerez : notre justice fait l'objet d'une défiance grandissante dont les causes sont en réalité multiples. Le projet de loi que je vous présente aujourd'hui vise précisément à inverser cette tendance qui altère notre démocratie et notre pacte social. Ce texte est d'abord le fruit de mon expérience d'avocat, qui m'a permis d'observer ce que notre justice faisait de meilleur, mais également de pire. Il est également le fruit du travail des commissions que j'ai installées dès mon arrivée à la chancellerie, mais également des commissions des lois des deux assemblées qui, monsieur le président Buffet, travaillent depuis de nombreuses années sur ces questions éminemment complexes.

Mais, à raison, les Français ne la comprennent plus, ne comprennent plus son langage, la trouvent tantôt trop sévère, tantôt trop laxiste et trop lente. Dans les jours qui viennent, nos débats devront répondre à certaines des attentes légitimes de nos concitoyens pour rendre la justice plus transparente, plus proche d'eux et plus protectrice de leurs droits en tant que justiciables.

En cinq ans, le budget de la justice aura augmenté de près de 33 %. Certes, nous partions de loin- un ancien garde des sceaux avait même évoqué la « clochardisation » de la justice mais qui pourrait nier l'implacable détermination du Président de la République, du Premier ministre et de ce gouvernement pour faire ce qui n'avait jamais été fait auparavant, à savoir donner à la justice de notre pays les moyens qu'elle mérite ? Parce que la défiance prospère souvent sur la méconnaissance, j'ai l'ambition de faire en sorte que tous nos concitoyens puissent mieux comprendre la justice du quotidien, celle qui est rendue dans les cours et les tribunaux de France en leur nom. Si les médias peuvent rendre compte des procès, ils ne peuvent pas filmer les audiences du quotidien. C'est tout l'objet de l'article 1 de ce projet de loi, qui apporte un changement d'importance. Je vous le dis d'emblée, je ne souhaite pas faire de la justice spectacle. C'est même tout le contraire C'est même tout le contraire : je veux que ces audiences filmées aient une vocation pédagogique, que notre justice soit enfin expliquée pour être mieux comprise. Le texte prévoit toutes les garanties pour assurer que la présence des caméras dans les prétoires ne porte pas atteinte aux droits des parties, tant lors de l'enregistrement que lors de la diffusion. Sans être exhaustif, je pense par exemple à l'autorisation d'enregistrement qui sera donnée par une autorité juridictionnelle et dans un motif d'intérêt public. garanties figurent encore dans la loi pour assurer la sérénité des débats, la présomption d'innocence, la sécurité des personnes, le droit à l'oubli, le respect de la vie privée, ou encore l'intérêt supérieur des mineurs ou des majeurs protégés. De même, la diffusion de l'audience ne pourra se faire qu'après une décision définitive. J'estime par ailleurs, depuis mes années d'avocature, que le lien de confiance qui est à reconstruire entre la justice et nos concitoyens repose aussi sur une meilleure connaissance mutuelle des professions du droit. C'est pourquoi j'ai souhaité expérimenter la participation d'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en tant qu'assesseur au sein des cours d'assises et des cours criminelles départementales. Aussi, je regrette que votre commission des lois ait supprimé ces dispositions novatrices. Dans le même esprit, j'ai souhaité que des magistrats président les commissions disciplinaires des avocats. Il est pour moi évident que la restauration de la confiance ne peut s'envisager sans le renforcement des droits auxquels les justiciables peuvent prétendre. À cette fin, j'ai souhaité que la durée des enquêtes préliminaires soit mieux encadrée et, donc, limitée dans le temps : les enquêtes de droit commun seront limitées à deux ans, avec la possibilité de les prolonger d'une année supplémentaire. Cette disposition restaure pleinement le rôle du ministère public en lui permettant non seulement de diriger les investigations, mais également de contrôler le rythme des enquêtes et, donc, de les traiter plus rapidement. un délai d'enquête dérogatoire porté à cinq années, et initialement réservé à la criminalité organisée et au terrorisme. Il me semble Il me semble nécessaire de le circonscrire aux infractions les plus complexes au risque de faire de l'exception la règle et, donc, une réforme pour rien Je suis donc défavorable à l'extension des dérogations voulue par votre commission, car elle viderait littéralement de leurs effets ces nouvelles dispositions. comme je l'avais déjà indiqué devant votre commission, et conformément à l'analyse du procureur national financier, je suis favorable, en matière économique et financière, à l'introduction d'une dérogation au régime d'enquête de droit commun, en la réservant aux seuls faits de corruption d'agents publics étrangers.

J'en viens maintenant à évoquer l'une des garanties les plus absolues du droit des justiciables, celle de la confidentialité de leurs échanges avec leur avocat. Je défends avec vigueur, dans ce projet de loi, le renforcement du secret professionnel des avocats, qui a trop longtemps été foulé aux pieds. Ce texte prévoit donc d'encadrer plus strictement les actes d'enquête comme les perquisitions, les écoutes téléphoniques ou l'exploitation des factures détaillées susceptibles de porter atteinte à cette confidentialité. J'ai entendu, comme vous, les craintes concernant l'efficacité des enquêtes, qui se trouverait soudainement mise à mal par le renforcement du secret professionnel des avocats. Dissipons ici les fausses querelles et les mauvaises caricatures Il est vrai qu'une enquête est toujours plus facile à conduire sans garanties pour les justiciables ou leurs avocats, mais nous sommes dans un État de droit

J'ajoute d'ailleurs que le problème n'est pas forcément bien posé : l'efficacité d'une enquête réside d'abord- nous y travaillons avec le ministre de l'intérieur -dans le nombre et la formation des enquêteurs spécialisés, notamment dans le domaine complexe de la délinquance économique et financière. Certains arguments que nous avons pu entendre à l'encontre du renforcement du secret professionnel témoignent d'une méfiance déplacée à l'encontre des avocats, alors qu'il s'agit- mais ai-je besoin d'en convaincre le Sénat ? -d'une profession fondamentale pour l'exercice des libertés et des droits démocratiques, et non d'un adjuvant de la délinquance. Si certains avocats commettent des infractions, la protection du secret professionnel ne trouve pas à s'appliquer. Enfin, il est faux, voire fantaisiste, de prétendre qu'il suffirait de mettre un avocat en copie de messages électroniques et de documents internes à une société

En cohérence, le Gouvernement émettra donc un avis de sagesse sur les amendements visant à rétablir cette disposition pour permettre, dans le cadre de la navette parlementaire, de trouver le meilleur des compromis. Parce qu'une justice qui inspire confiance est aussi une justice rapide, qui ne correctionnalise pas les affaires de viol, je crois qu'il est absolument indispensable de maintenir dans le texte la généralisation des cours criminelles départementales.

les débats à venir vont nous permettre de travailler ensemble au remplacement du rappel à la loi. Cette alternative aux poursuites était devenue incompréhensible pour nos concitoyens, ainsi que pour les forces de l'ordre qui la mettaient en oeuvre. Pis, elle portait gravement atteinte à l'autorité de l'État. C'est pourquoi je vous proposerai la création d'un « avertissement pénal probatoire », élaboré en concertation avec les magistrats de terrain, la conférence nationale des procureurs de la République, afin d'apporter une réponse pénale plus lisible et plus efficace. Pour faire simple, lorsqu'un justiciable se verra remettre cet avertissement pénal probatoire, on lui rappellera ses obligations légales sans le poursuivre. En revanche, si dans l'année qui suit, il commet une nouvelle infraction, on ressortira son dossier et on le poursuivra au titre de la nouvelle infraction- cela va de soi -, mais aussi de l'ancienne. Afin d'éviter les écueils précédents, cette mesure ne pourra être prononcée que si la personne a reconnu sa culpabilité et n'a pas déjà été condamnée. Elle ne pourra pas non plus s'appliquer aux cas de violences et de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Enfin, la solennité de cette nouvelle réponse pénale sera renforcée, car seul un procureur ou son délégué pourra la prononcer. Je précise que, afin de préparer le transfert de charges entre services enquêteurs et autorités judiciaires, cette nouvelle disposition n'entrera en vigueur que progressivement. Avoir confiance en la justice, c'est aussi comprendre le sens de la peine et surtout la manière dont elle est exécutée. Pour cela, il est devenu indispensable de refondre entièrement le dispositif des réductions de peine, pour le rendre d'abord plus compréhensible, mais surtout plus juste. Il convenait d'abord d'en abroger le caractère automatique. Je souhaite que, désormais, les réductions de peine soient graduées au mérite et que la personne détenue sache enfin clairement ce qui est attendu d'elle en termes de conduite et d'efforts de réinsertion. c'est bien sur ces deux aspects que l'autorité judiciaire se prononcera pour envisager ces réductions, notamment à partir de l'avis des personnels pénitentiaires. Mais mieux prévenir de nouveaux passages à l'acte passe également par la réduction des sorties « sèches C'est dans cette optique que sera créée une libération sous contrainte, avec un accompagnement à trois mois de la fin de la peine. Il ne s'agit évidemment pas d'une mesure de faveur, mais bien du prolongement de l'exécution de la peine de la peine prononcée, sous d'autres modalités, afin de favoriser, dans l'intérêt de la société, la réinsertion du condamné. C'est dans cette même logique de renforcement de la réinsertion que je soutiens la création d'un contrat de travail pour le détenu. En se rapprochant du droit commun, ce contrat permettra de mieux préparer les personnes détenues, souvent dépourvues de toute expérience professionnelle, à retrouver une place dans la société. Il permettra également de revaloriser l'image du travail pénitentiaire à l'extérieur et d'attirer les entreprises qui veulent s'inscrire de responsabilité sociétale. Je précise, parce que je connais vos inquiétudes, madame, monsieur les rapporteurs, que je peux d'ores et déjà prendre l'engagement devant vous que les coûts liés à ces nouveaux droits seront pris en charge par l'État et qu'ils ne seront pas supportés par les entreprises qui feront le choix louable d'intervenir en prison. Enfin, le lien de confiance que nous souhaitons retisser entre nos concitoyens et leur justice ne peut être conçu sans une discipline renforcée et rénovée des professions du droit, sans replacer l'usager au centre du dispositif. Ce dernier sera désormais assuré que chacune de ses réclamations sera traitée avec célérité et impartialité. Je me félicite que cette réforme importante et largement consensuelle ait pu se construire avec les professions, mais aussi que votre commission l'ait sensiblement enrichie. Toujours pour répondre aux attentes des usagers, le texte comporte des dispositions modernisant les conditions de fonctionnement de la justice. En particulier, il prévoit toute une série de mesures pour encourager le recours aux modes amiables de règlement des différends,

Afin de satisfaire les besoins concrets exprimés par les justiciables, je vous proposerai également de faciliter le recours à la visioconférence, à la demande des parties, pour tenir des audiences en matière civile et commerciale. Comme je m'y étais solennellement engagé devant l'Assemblée nationale, je vous proposerai d'enrichir ce texte d'un nouvel article visant à créer un conseil de l'accès au droit sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, où l'absence d'une telle structure n'est plus tolérable. Il s'agit, dans la droite ligne de la justice de proximité que je défends, de permettre le développement du réseau d'accès au droit avec l'appui des juridictions, professions du droit, provinces, maires, autorités coutumières et monde associatif. Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, de changer le regard de nos compatriotes sur l'institution judiciaire. Bien sûr, un projet de loi ne résoudra jamais à lui tout le problème de la défiance des Français envers leur justice, mais ses dispositions portent toutes en elles de quoi susciter un choc de confiance qu'il nous appartiendra de de prolonger lors des États généraux qui s'ouvriront prochainement. Sans tabou ni censure, nous continuerons à y travailler avec passion.

sixième réforme de la justice depuis le début du quinquennat, annonce clairement son ambition : redonner confiance dans la justice. Ambition d'autant plus forte que plus d'un Français sur deux- très exactement 53 % -ne croit pas en la capacité de la justice à répondre à ses attentes : une justice de qualité, simple dans son fonctionnement, rapide dans ses décisions et effective dans l'exécution de ses jugements. Cette inquiétude, le Sénat la partage ! C'est pourquoi nous avons formulé de nombreuses propositions pour le redressement de la justice, clé de la confiance de nos concitoyens dans l'institution judiciaire. Cette ambition, nous continuons à l'alimenter par nos propositions issues de l'Agora de la justice, qui s'est tenue hier et qui a permis des échanges éclairants. C'est dans ce même état d'esprit que mon collègue rapporteur Philippe Bonnecarrère et moi-même avons mené nos travaux sur ce texte qui affiche une ambition volontaire, mais qui est malheureusement avant avant tout un catalogue de mesures souvent très techniques et de portée inégale. En effet, monsieur le garde des sceaux, la confiance ne se décrète pas : elle s'acquiert ! Et pour ce faire, il convient d'en assurer les conditions,

Aussi, afin d'éviter les dérives et d'assurer la transparence recherchée, nous avons précisé que leur objectif doit être « pédagogique, informatif, scientifique et culturel », et que la participation des parties au procès ainsi diffusé Pour rétablir cette confiance, il semble avant tout urgent d'apaiser le monde judiciaire : magistrats, avocats, policiers, greffiers et officiers publics, tous ceux qui, par leur engagement quotidien, font vivre la justice, mais qui sont trop souvent la cible d'attaques infondées. des sceaux, que l'augmentation, ces deux dernières années, des crédits de votre ministère ait permis de renforcer les moyens humains tant attendus. Mais c'était sans compter l'accumulation de réformes législatives qui se sont avérées difficilement assimilables dans des délais rapprochés et qui déstabilisent l'institution judiciaire. La généralisation des cours criminelles départementales nous semble tout aussi précipitée. Lancée en 2019, l'expérimentation doit se prolonger jusqu'en mai 2022 et se conclure par la remise d'un rapport au Parlement. Si les premiers retours semblent positifs, force est de constater qu'ils ne portent que sur un nombre restreint d'affaires, perturbées par la crise sanitaire et la grève des avocats. Faute de recul suffisant, nous avons décidé de prolonger cette expérimentation jusqu'au mois de mai 2023. Toujours dans un souci d'apaisement et de clarification du rôle de chacun, la commission a supprimé la présence des avocats honoraires dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Le contrat d'emploi pénitentiaire, qui n'est pas un contrat de travail, mais se rapproche du droit du travail, constitue ainsi une avancée sociale en créant un lien direct entre le détenu et son employeur. Cependant, nous serons vigilants à ce que des règles trop contraignantes et un coût du travail augmenté ne découragent pas les opérateurs économiques et à ce que ce coût soit réellement supporté par l'État. Enfin, dévoilé tardivement, l'avertissement pénal probatoire, annoncé après la suppression du rappel à la loi, offrira une alternative nécessaire aux poursuites, ciblée sur les infractions les moins graves émanant de primodélinquants. Victor Hugo affirmait : « Faire justice est bien, rendre justice est mieux. » C'est en nous appuyant sur les professionnels de la justice que nous reconstituerons collectivement le lien entre les Français et l'institution judiciaire, base de notre État de droit.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat aborde la discussion de ce texte de manière constructive.

ils ont l'avantage d'être connus, assumés et argumentés de part et d'autre, ce qui devrait permettre, monsieur le garde des sceaux, une décision mûrie dans un bicamérisme de bon aloi.

un autre texte, sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, tandis que nos magistrats se préparent à en appliquer dans quelques jours un troisième, issu d'une ordonnance

pourrait se dire qu'elle est en train de refaire surface, pour les uns, ou d'entamer sa remontée, pour les autres, vous proposez de nouveaux objectifs, de nouvelles procédures, de nouvelles dépenses ! Voilà, vraiment, provoque notre étonnement, ce que je qualifie de paradoxe : il va y avoir de nouveaux délais à surveiller, de nouvelles procédures à mener, qui vont nécessiter plus de juges d'instruction et de juges de l'application des peines, il va y avoir des ordonnances supplémentaires à motiver, des complexités de procédure supplémentaires, voire dépenses de fonctionnement pures et dures, comme celles que vous venez d'annoncer, il y a quelques minutes, quant à la prise en charge des cotisations sociales des employeurs dans le cadre du nouveau régime

Sans une justice forte et efficace, c'est l'ensemble de la société qui vacille. Nous avons été nombreux à rappeler que la moitié des Français n'ont plus confiance en notre justice. Ces chiffres sont des alarmes auxquelles il est urgent de répondre. Le premier problème de la justice, c'est celui des moyens. À cet égard, je veux saluer l'action du garde des sceaux, qui a obtenu pour 2021 une augmentation de budget significative. Nous souhaitons que l'effort soit poursuivi pour les années à venir. Nous y serons attentifs lors de l'examen du prochain projet de loi de finances. Cependant, pour que la justice cesse d'être le coupable idéal, il est également nécessaire de mieux faire connaître son fonctionnement. Nous sommes donc tout à fait favorables à la diffusion des procès pour des motifs d'intérêt général. Nos deux rapporteurs, dont je salue le travail, ont apporté des précisions utiles quant aux modalités de ces diffusions. Nous espérons que cette mesure permettra au plus grand nombre de comprendre ce que les jurés savent bien : juger en connaissance de cause n'est jamais facile. La justice a besoin de transparence quand elle est rendue ; elle a besoin de secret quand elle se prépare. Nous soutenons donc le renforcement des sanctions en cas de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction. Il est essentiel de préserver ces secrets jusqu'à ce que les investigations soient terminées. Nous voyons trop souvent des condamnations morales tomber dans la presse alors que le verdict n'est pas encore rendu par les juges. Cela n'est pas acceptable. Par essence, la phase d'enquête ne peut être que temporaire. La limitation de la durée des enquêtes préliminaires est une très bonne mesure. Il faudra néanmoins s'assurer que les moyens humains des services d'enquête permettront de respecter ces délais sans que la qualité du travail en pâtisse. Le même souci d'efficacité doit guider la phase de jugement. Concernant certains crimes, notamment les crimes sexuels, notre commission des lois a souhaité prolonger l'expérimentation des cours criminelles plutôt que la pérenniser. Cette décision de prudence ne remet pas en cause les résultats satisfaisants que l'expérimentation a produits. Il est essentiel que ces crimes reçoivent une réponse pénale forte. La justice de notre pays doit remplir un double objectif d'équité et de fermeté, pour que les citoyens retrouvent confiance en elle. À cet égard, notre groupe soutient particulièrement la suppression des réductions de peine automatiques. Le manque de places de prison ne peut motiver ce dispositif qui envoie un message délétère, car seul le bon comportement du détenu doit justifier une réduction de peine. Il faut récompenser celui qui renoue avec les valeurs de notre société et qui prépare ainsi sa réinsertion. Cette mesure nécessite cependant que le nombre de places de prison soit augmenté en conséquence. Dans la même optique de réinsertion, nous voulons saluer l'encadrement du travail des détenus par un contrat d'emploi pénitentiaire. « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin », disait Voltaire. Ce qui se trouve au fondement de notre société ne doit pas s'arrêter aux portes de la détention. C'est par le travail que l'individu s'améliore : il est donc encore plus nécessaire que les détenus y aient accès. traitent encore beaucoup d'autres points que je ne pourrai évoquer par manque de temps. Je constate cependant que ces textes n'abordent que peu la justice civile et commerciale, qui constitue pourtant l'une des principales voies d'accès des Français à la justice. Néanmoins, je relève qu'il y est prévu de permettre l'apposition de la formule exécutoire sur l'acte d'avocat issu d'un mode alternatif de règlement des différends. J'y suis favorable, dans la mesure où cette disposition incite à recourir à ces modes qui désengorgent nos tribunaux, tout en sécurisant l'accord trouvé par les parties. Les dispositions contenues dans ces textes sont porteuses de progrès pour notre justice. Pour que les Français retrouvent confiance en elle, il est essentiel de renforcer sa publicité, de clarifier et d'affermir les sanctions. Notre groupe soutiendra donc leur adoption, tout en insistant sur la nécessité de lui donner les moyens de remplir ses missions.

voici face à un texte qui nous laisse un vrai goût d'inachevé, de « presque », de « juste à côté ». L'intention est louable. Le constat d'une justice trop incomprise et éloignée des Français la réponse à la lenteur et aux difficultés de la justice ne doit pas uniquement consister à rogner sur les droits de la défense, sur l'initiative des magistrats enquêteurs, sur la capacité du juge à juger. En entamant la lecture de ce projet de loi, je le regardais comme ce qu'il est : une réflexion qui devrait couronner une fin de mandat en matière de justice. Mais, une fois ce texte ficelé, à la fois par la commission des lois et par le Gouvernement, la morale que j'en retiens serait plutôt celle-ci : la justice est trop lente, court-circuitons la justice ! Certes, le constat d'une justice trop lente et perdant de son efficacité est partagé par tous, mais quels remèdes y apportez-vous ? Dans la course à l'amélioration des chiffres et à l'affichage,

Que dire des transferts de tâches entre professionnels du droit ! À vouloir afficher un changement radical, vous ne permettez d'améliorer profondément ni les conditions d'accès à la justice ni les conditions de travail des magistrats.

je me demande même si certains ne rêveraient pas de remplacer les humains par des machines ou des algorithmes à juger ! Je regrette également de ne rien voir sur la justice des mineurs, dont vous savez qu'elle est en souffrance : des délais trop longs, des prises en charge inadaptées- et pourtant, rien ! Ah, si

sert essentiellement à apporter de l'eau au moulin de ceux qui affirment que la justice ne condamne pas assez. De manière générale, aucune des mesures de ce texte qui touchent à l'exécution des peines ne découle d'une réflexion profonde rien sur le développement des travaux d'intérêt général. La prison n'est pas, n'en déplaise à certains, la seule sanction efficace dans notre arsenal : encore faut-il juger l'efficacité d'une sanction Cette ambition de sanctionner toujours plus fort, forcément par de la prison, ne s'accompagne pourtant d'aucun apport sur les conditions de vie des détenus. Je ne saurais trop rappeler les condamnations répétées de notre pays pour des conditions de détention proches de l'indignité, comme l'a récemment souligné la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté au sujet des lieux de garde à vue.

là nous paraît non seulement manquer de vision globale, mais surtout marquer une dérive vers une justice de plus en plus punitive et vindicative, dont le seul but serait d'emprisonner les gens au plus vite et le plus longtemps possible. Certes, cela répond à une demande de fermeté accrue, mais nous ne sommes pas dupes : il s'agit d'un leurre dont rien ne démontre l'efficacité. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre ce texte.

le colloque organisé hier soir par notre commission des lois l'a confirmé, notamment au moyen des résultats d'une enquête d'opinion présentés à cette occasion : nos concitoyens accordent à notre institution judiciaire une confiance et un crédit limités. Ce constat doit être considéré, déjà, pour ce qu'il exprime du rapport complexe, voire conflictuel, d'une partie non négligeable de la population à des institutions indispensables au fonctionnement de notre société. aussi parce que, comme nous l'avons constaté hier, il heurte les acteurs de cette institution, dont la réalité de la pratique et des décisions, réalité elle aussi chiffrée par des données malheureusement moins exploitées dans le débat public et médiatique, diverge du sentiment et de l'impression dégradés qu'on ressent envers la justice. Ce décalage doit lui aussi être traité, nous en conviendrons tous. Il doit l'être non pas pour livrer la justice au tribunal de l'opinion, ou encore pour légiférer dans le seul but d'infléchir la sentence de celui-ci, Bas l'a d'ailleurs bien exprimé hier, mais pour saisir les ressorts de la défiance et agir sur ceux-ci lorsqu'ils procèdent bien de mécanismes qui ne fonctionnent pas, ou plus assez bien. il a été rappelé, plusieurs causes rationnelles peuvent être invoquées à l'appui du constat précité : la lenteur de certaines procédures, la méconnaissance du fonctionnement de la justice- opaque pour 69 % des Français -, ou encore l'enjeu du sens de la peine. Au-delà de cet état des lieux, sur lequel nous pouvons nous accorder, se pose bien sûr la question des solutions à apporter, des voies à emprunter pour y répondre avec pertinence et efficacité. On peut certes, comme le font certains de nos collègues aujourd'hui, appréhender le projet de loi soumis à notre discussion en creux, par ses manques. D'ailleurs, s'attacher à souligner ce que ce texte n'est pas peut aussi, à rebours de certains positionnements, nous amener à souligner les autres vecteurs de confiance mobilisés par le Gouvernement, qu'il s'agisse de la justice de proximité, de la hausse importante des moyens- condition de toute réforme ambitieuse -ou encore des prochains États généraux de la justice, qui s'inscriront sans doute dans l'esprit constructif de l'Agora d'hier soir. Mes chers collègues, si l'on se concentre à l'inverse sur le fond du présent projet de loi, force est de constater qu'une convergence se dessine sur l'esprit de ce texte et sur la majorité de ses dispositions. C'est le cas s'agissant de la nécessité, pour mieux faire connaître le fonctionnement de l'institution judiciaire, d'ouvrir les possibilités d'enregistrement et de diffusion des audiences, sous réserve bien sûr de garanties, dont certaines ont été utilement renforcées par nos rapporteurs. Un consensus se dessine également quant à la nécessité, pour renforcer les droits des justiciables, d'ouvrir les enquêtes préliminaires au principe du contradictoire et de les encadrer dans le temps, ménageant des exceptions pour tenir compte de la complexité de certaines enquêtes en matière de délinquance économique et financière. Le bon curseur du champ d'application de l'allongement dérogatoire de la durée de l'enquête pourra continuer à nourrir nos échanges, mais il me semble qu'un souci d'équilibre nous réunit. L'un des L'un des facteurs de la confiance réside également dans le respect des droits de la défense, qui répond non à une lubie corporatiste, mais bien à une volonté de protection des justiciables et de leur présomption d'innocence. À ce titre, le renforcement de la protection du secret de l'enquête et de l'instruction a été utilement conforté par nos rapporteurs. Les dispositions relatives à la révision et à l'harmonisation de la déontologie et de la discipline des professions du droit, améliorées de manière substantielle en commission, sont elles aussi de nature à intégrer l'enjeu de la protection des droits de ceux qui y ont recours et, là aussi, à offrir l'égalité des armes. La confiance dans l'institution judiciaire est indissociable, enfin, du sens de la peine, de la réinsertion des personnes condamnées et de la prévention de la récidive, mais également de la compréhension de la réponse pénale par l'ensemble des justiciables. Dans le sens de la peine, c'est finalement la préservation de la sécurité de notre société qui est en jeu, dépassant toute polarisation ou toute cristallisation des oppositions politiques. Je veux à ce titre souligner plusieurs dispositions du présent projet de loi : la systématisation de la libération sous contrainte en fin de peine pour les infractions de basse intensité, afin d'éviter les sorties dites la suppression de l'automaticité des crédits de réduction de peine, car l'effort a également sa place dans le sens de la peine ; enfin, le contrat d'emploi pénitentiaire, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des personnes condamnées. Sur la plupart de ces dispositions, là encore, une convergence se dessine sur nos travées. Le remplacement du rappel à la loi par un avertissement pénal probatoire s'inscrit dans cette finalité de confortement du sens, par un renforcement du caractère solennel et de la compréhension de la mesure. Il faut bien rappeler que la solution proposée se distingue réellement du rappel à la loi ; elle rejoint d'ailleurs la rédaction initialement envisagée par nos rapporteurs, en ce qu'elle impose l'intervention du procureur de la République ou de son délégué, ainsi que la réparation du préjudice causé à la personne morale ou physique, et qu'elle comporte une période probatoire. Mes chers collègues, certains points nourriront nos débats dans les prochaines heures. Je pense notamment à la présence de l'avocat lors des perquisitions, ou encore à la mise en balance de l'opportunité d'un allongement d'un an de l'expérimentation des cours criminelles avec celle de leur généralisation immédiate. Les différentes dispositions qui nous réunissent ce soir rappellent en tout cas à quel point la confiance des justiciables, mais aussi des acteurs de la justice, en la capacité de cette dernière à remplir son office est indissociable de notre pacte social,

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, comment restaurer la confiance dans la justice quand près de la moitié de la population n'y croit plus ? Voilà la question qui nous est posée au travers de ce projet de loi. Ce constat, posé par nombre de nos concitoyens, est tout aussi criant qu'il est contradictoire : en cela il est typiquement français ! Il est contradictoire, car les Français sont partagés entre, d'une part, les tenants du tout répressif, du tout carcéral- ou, du moins, du très répressif -et, d'autre part, ceux qui pensent que cette solution ne fonctionne plus et qu'il nous faut davantage nous orienter vers des peines alternatives, qu'il faut vider les prisons plutôt qu'en construire de nouvelles. Je grossis volontairement le trait, mais je partage largement cette seconde approche, notamment dans un domaine que je connais, celui de la protection judiciaire de la jeunesse, où, pour de nombreux jeunes, l'incarcération en centre éducatif fermé est le premier pas vers la récidive et le début d'un parcours judiciaire tortueux. Au-delà de ces débats, les Français sont tous d'accord sur un point : entre la commission d'une infraction, le prononcé d'une peine et son exécution s'écoule souvent beaucoup trop de temps. La France a par ailleurs été condamnée de nombreuses fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce manque de célérité. Vous me permettrez d'émettre quelques regrets avant d'en venir au texte. Tout d'abord, ce texte ne comporte pas ou peu de dispositions concernant la justice du quotidien qu'est la justice civile.

preuve une nouvelle fois que, si la justice civile est omniprésente dans la vie de la société, elle demeure invisible dans le débat public. À cela s'ajoute l'impression que ce texte est un peu décalé, alors que les États généraux de la justice, annoncés depuis de nombreux mois, sont sur le point de débuter. Malgré ces manques évidents et un calendrier contraint, la commission des lois a apporté quelques modifications substantielles au texte initial qui peuvent, pour partie, C'est le cas de l'article 1 portant sur l'enregistrement et la diffusion des audiences : la commission des lois a apporté davantage de garanties en précisant la nature du motif d'intérêt public, en évitant toute possibilité de rémunération pour les personnes enregistrées

nous partageons la volonté de la commission des lois de prolonger l'expérimentation avant sa généralisation, afin d'avoir davantage de recul sur ce dispositif. Sur le sujet de la concurrence entre les cours criminelles et les cours d'assises, si vous vous vous vous êtes voulu rassurant, monsieur le garde des sceaux, je me permets de vous rappeler notre attachement et celui de nombreux Français aux assises, qui restent le dernier lien direct entre eux et leur justice.

Lors de l'examen de ce texte, nous serons vigilants au sort réservé à nos différents amendements, notamment sur la médiation ou sur les mesures concernant les huissiers de justice. Restent deux interrogations. interrogation concerne le remplacement du rappel à la loi par l'avertissement pénal probatoire. Si nous sommes plutôt favorables au principe de cette mesure, nous regrettons que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une étude d'impact qui nous aurait très certainement éclairés.

que l'enquête porte sur un contentieux fiscal ou un délit financier : cela porte atteinte à l'exercice professionnel de l'avocat. Pour conclure, il convient de souligner, pour le saluer,

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis nous laisse, comme d'autres, pour le moins sceptiques sur la forme comme sur le fond. le fond. Nous nous interrogeons également sur le contexte dans lequel intervient un tel débat. Il semblerait en effet que, à la veille d'échéances électorales importantes, les projets, débats, états généraux en tout genre sur le thème de la justice, surgissent de toutes parts,

Certes, filmer les audiences pourrait présenter une vertu pédagogique en donnant aux justiciables accès aux rouages de la justice du quotidien- nous n'y sommes pas opposés, à condition d'encadrer sérieusement ce dispositif -, mais bien d'autres problématiques amputent aujourd'hui la confiance de nos concitoyens dans cette institution. Il est par exemple important de faire le constat amer des suspicions de nos concitoyens quant à l'impartialité des juges et à leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Bien plus, nous ne pouvons ignorer l'impact notable de l'indigence des moyens de la justice sur la qualité des audiences et de la motivation, sur les délais d'audiencement et de jugement- autant d'éléments qui ont une incidence non négligeable sur la mauvaise opinion que les citoyens peuvent se faire de leur justice, et ce malgré l'engagement de l'ensemble des professionnels pour faire mieux au quotidien. Toutes ces questions ne sauraient donc être résolues par la simple diffusion d'images d'audience à la télévision ou sur internet : elles nécessitent des réformes institutionnelles permettant de renforcer dans les faits le statut des magistrats- la réforme sur l'indépendance du parquet est-elle définitivement enterrée ? -ou encore d'encadrer les transmissions d'informations des juridictions à la Chancellerie. Permettez-moi une digression : nous avons vu qu'il ne suffisait pas d'organiser des débats télévisés avec de grands professeurs de médecine pour rassurer nos concitoyens sur les politiques sanitaires à conduire. Enfin, ce projet de loi qui affiche l'ambition de renouer le lien de confiance entre justiciables et institution judiciaire manque cruellement de crédibilité en éludant la question de la justice civile, au coeur du quotidien de nos concitoyens. contient une seule disposition, minime, mais néanmoins positive, la suppression de la juridiction nationale des injonctions de payer, bien que cela n'aille pas du tout dans le sens d'une confiance renforcée dans la politique menée par le Gouvernement en matière de justice, le garde des sceaux actuel supprimant une juridiction créée par la garde des sceaux qui cours de ce quinquennat. Venons-en à ce que le texte contient de positif. Nous saluons les mesures concernant le travail en détention. Le contrat d'emploi pénitentiaire marque indubitablement un progrès ; il consacre des relations entre les donneurs d'ordre et le travailleur détenu. le Gouvernement demande l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnances. Concernant l'exécution des peines, alors qu'un pas est fait dans le sens de la régulation carcérale en rendant automatique la libération sous contrainte à trois mois de la fin de peine, ce qui est donné, d'un côté, est repris de l'autre, avec la fin des crédits de peine attribués d'emblée lors du placement sous écrou des détenus. Nous y reviendrons lors de la articles. En l'état, ce projet de loi ne peut recueillir notre assentiment. Si un certain nombre de mesures semblent plutôt positives, par exemple celles qui visent à encadrer le travail en détention ou encore celles qui sont relatives à l'évolution des règles déontologiques et disciplinaires des professionnels du droit, d'autres sont pour nous rédhibitoires, rédhibitoires, à l'instar de la fin des crédits de réduction des peine, de la suppression du rappel à la loi, finalement remplacé par ce qui pourrait s'apparenter à un Canada Dry de la justice, ou encore de la généralisation des cours criminelles départementales. Les crimes sexuels ne peuvent être jugés au rabais et à la place du peuple à travers les jurés populaires ; la cour d'assises doit rester centrale dans le fonctionnement de la justice. Dans l'ensemble, trop de mesures vont dans le sens d'une gestion

dans tout pays démocratique, l'État de droit se mesure à l'aune de l'adhésion et de la confiance qui lient les citoyens et les institutions régaliennes. Force est de constater que, dans notre pays, si la confiance à l'égard de l'armée, de la gendarmerie et de la police est élevée, celle que les Français placent en la justice est altérée, parfois même dégradée. En effet, dans une enquête d'opinion de 2019, un Français sur deux signifiait sa défiance à l'égard de notre système judiciaire judiciaire et 62 % des Français indiquaient que la justice fonctionnait mal. Ces chiffres sont durs, ils sont même cruels à bien des égards, car ils témoignent d'un décrochage profond entre les Français et l'institution judiciaire. Les causes de cette défiance sont à la fois multiples et justifiées. Nos tribunaux sont engorgés, les magistrats et les greffiers croulent sous les dossiers. Deux exemples très récents : au tribunal judiciaire de Nîmes, il n'y a plus de juge d'instruction spécialisé en matière économique et financière

les inégalités territoriales dans l'accès à la justice sont criantes. Les procédures rallongent les délais de traitement et d'audiencement. De surcroît, en dépit du travail sérieux qu'accomplissent les associations d'aide aux victimes, les parties civiles ont le sentiment d'être oubliées, voire délaissées. Certaines victimes apprennent par exemple que leur plainte a été classée sans suite, sans que personne ait pris le soin de les en informer. Monsieur le garde des sceaux, lors de votre prise de fonction, vous avez annoncé vouloir « améliorer la justice dans notre pays regrettant alors « les conditions de travail déplorables dans lesquelles se débattent quotidiennement magistrats et greffiers » et estimant nécessaire de mettre en place une justice plus proche du citoyen. Pour l'heure, votre bilan est pour le moins contrasté : l'augmentation bien réelle des crédits qui vous ont été accordés lors du vote du précédent projet de loi de finances reste cependant insuffisante pour corriger les nombreux travers d'un système judiciaire laissé exsangue. Indépendamment de la question des moyens, qui est centrale, il y a le contexte dans lequel nous sommes invités à débattre de ce projet de loi. Il règne objectivement un climat de perplexité, voire de crispation, chez les acteurs du système judiciaire, qui ont été déçus par le contenu de ce projet de loi. Derrière un titre ambitieux qui aurait pu séduire et qui aurait dû convaincre, il n'y a qu'une addition de mesures techniques et quelques ajustements qui évitent soigneusement les vrais problèmes et ne règlent en rien la justice du quotidien. Je relève enfin que nous sommes saisis de ce projet de loi alors même que le Gouvernement annonce son intention d'organiser des États généraux de la justice. Cette multiplication d'annonces vient brouiller le message gouvernemental et ne favorise pas les conditions de la confiance. Monsieur le garde des sceaux, la confiance dans l'institution judiciaire ne se proclame pas, pas plus qu'elle ne se décrète. La confiance dans l'institution judiciaire se construit jour après jour, elle se mérite. Venons-en au contenu de votre projet de loi. Sans nier l'intérêt pédagogique que peuvent représenter la captation vidéo des audiences et leur retransmission à la télévision, nous avons du mal à évaluer l'impact réel d'une telle mesure sur la confiance des Français dans l'institution judiciaire. Plus surprenant encore, alors que vous sembliez, comme nous, attaché aux jurys populaires nés de la Révolution française, vous voulez désormais supprimer les cours d'assises et les remplacer par les cours criminelles départementales. En 2017, sur France 3 Corse, vous critiquiez vous critiquiez les cours criminelles départementales, indiquant que la présence des citoyens était une « bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges Et d'ajouter : « La justice est rendue au nom du peuple et on voudrait interdire au peuple de rendre justice ? Nous avons besoin du jury populaire ; moi, je ne veux pas d'une justice qui soit exclusivement professionnelle. » Monsieur le garde des sceaux, vous avez parfaitement le droit de changer d'avis, vous avez même le droit d'évoluer, mais avouez qu'il y a quelque paradoxe à évincer les Français quand ils sont acteurs de la justice, notamment lorsqu'ils siègent dans les cours d'assises, pour les réduire au simple statut de téléspectateurs devant une émission à mi-chemin entre et. Très bien ! La réforme des

Pour autant, l'ensemble des professionnels que nous avons rencontrés et auditionnés soutiennent qu'il n'y a pas lieu de légiférer sur cette question et que la nouvelle réforme pourrait avoir deux effets pervers majeurs. D'une part, elle engendrera la multiplication des sorties « sèches », entravant ainsi la volonté gouvernementale, que nous partageons, de lutter contre les récidives puisque le détenu ne pourra pas pleinement préparer sa réinsertion dans la société.

rappels à la loi en 2019. Monsieur le garde des sceaux, supprimer un rappel à la loi et ne le remplacer par aucune mesure alternative, c'était le meilleur moyen d'accréditer involontairement, je vous l'accorde, ce sentiment d'impunité judiciaire chez certains auteurs d'infractions. Supprimer le rappel à la loi et ne le remplacer par aucune mesure alternative, c'était prendre le risque de faire plonger les statistiques en matière de réponse pénale. C'est faux ! En effet, je souligne, pour mémoire, que les rappels à la loi représentent la moitié des mesures alternatives aux poursuites. Vous vous êtes ravisé et c'est tant mieux. N'en déplaise à ses détracteurs, le rappel à la loi a prouvé sa vertu dissuasive en vingt ans de pratique. Aux incohérences de fond que contient ce projet de loi s'ajoute la forme choisie pour en traiter certains aspects essentiels le groupe socialiste déplore que le Gouvernement ait initialement choisi d'avoir recours aux ordonnances pour les articles 14, 15, 27 et 32. Monsieur le garde des sceaux, il appartient au Parlement de légiférer. L'usage abusif que fait de l'article 38 de la Constitution depuis le début de cette législature n'est pas acceptable. Le recours trop fréquent aux ordonnances et à la procédure accélérée n'est pas respectueux du Parlement et des parlementaires.

La commission des lois a partiellement satisfait cette demande et je souhaite en profiter pour remercier les rapporteurs de la qualité de leur travail. Pour espérer obtenir et gagner la confiance des Français, le préalable consisterait peut-être à jeter les bases d'un travail loyal, respectueux et constructif avec les parlementaires que nous sommes,

n'est proposé en matière de justice civile, commerciale et familiale ; or le contentieux civil totalise 2,2 millions de décisions rendues par an, quand la justice pénale n'en rend que 800 000. Il est grand temps que nous nous penchions sur cette justice du quotidien, celle qui a un impact sur nos concitoyens.

Pour éloigner ce funeste destin, notre groupe s'attachera à gommer les imperfections de ce texte et à lui donner un peu plus de consistance lorsque c'est nécessaire. Nous espérons que vous saurez accueillir nos propositions avec ouverture ; cela est d'autant plus souhaitable que, dans cet hémicycle, nous sommes, les uns et les

dès l'abord, je dois vous dire que j'ai été un peu surpris du décalage entre le titre, l'objet annoncé de ce texte et son contenu réel.

le caractère quelque peu présomptueux de l'intention affichée par ce texte. J'espère néanmoins que nos travaux contribueront à ce qu'un certain nombre de dispositions utiles s'intègrent à notre corpus juridique. Toujours est-il que, entre le déroulement de l'enquête préliminaire, l'adaptation du régime des droits de la défense, les cours criminelles, la possibilité de filmer l'audience, le recours à des magistrats non professionnels, nous ne sommes tout de même pas dans un Grand Soir du service public de la justice. D'ailleurs, le texte paraît déjà incomplet, puisque le Gouvernement en annonce d'autres, comme s'il avait tant de temps devant lui pour faire en quelques mois ce qui n'aurait pas été fait en cinq ans. Il serait donc plus exact et moins présomptueux d'intituler ce texte « projet de loi portant diverses dispositions relatives à la justice ». Ce ne serait déjà pas si mal et cela renseignerait davantage le public sur son contenu réel. En réalité, monsieur le garde des sceaux, convenons-en, cette question est tout à fait secondaire le titre du texte sera bien vite oublié sous l'effet de la codification. Je crains d'ailleurs que son contenu ne le soit à son tour assez rapidement aussi. vous avez souhaité organiser des États généraux de la justice. Nous nous sommes mis en situation d'y prendre part. L'Agora de la justice,

face à l'énoncé des différents points de vue exprimés par les Français sur la justice, il y avait dans le corps des magistrats, mais aussi chez les avocats, les responsables de l'administration pénitentiaire, voire les universitaires, beaucoup d'émotion, ce qui nous a permis de mesurer de nouveau à quel point tous ceux qui concourent à la justice sont sincèrement et profondément engagés pour le bon fonctionnement de ce grand service public. Nous voulons aider la Chancellerie à renouer avec la communauté judiciaire en même temps qu'à resserrer les liens distendus entre les Français et la justice. Je crois, après vous avoir entendu, monsieur le garde des sceaux, que vous partagez largement ce constat pourtant sévère. Reste que je préfère un garde des sceaux objectif sur la situation dont il a la responsabilité à des discours de marchand de bonheur qui ne devraient pas avoir cours en ce qui concerne la justice. vous avez raison sur un point essentiel : on ne peut laisser perdurer la défiance que mesurent les enquêtes d'opinion entre les Français et la justice ni laisser la justice livrée en pâture au tribunal de l'opinion. Je le dis au Gouvernement : les États généraux doivent commencer par un état des lieux, lequel, s'il veut servir à un débat consensuel entre les Français, doit être loyalement établi, objectif et impartial. Il y a la justice civile : plus de 2 millions de décisions sont rendues chaque année ; ces décisions concernent la famille, la consommation, les loyers, mais aussi, avec la justice prud'homale, les licenciements ou les salaires. Ces décisions touchent le quotidien des Français. Il n'en est pas question dans ce texte. Pourtant, rares sont nos concitoyens qui n'ont pas au moins une fois dans leur vie besoin de l'arbitrage d'un Ce n'est donc pas accessoire. Hélas, après cinq années du quinquennat actuel, nous constatons que les délais moyens de jugement ne se sont pas raccourcis : ils se sont au contraire encore allongés d'un mois, pour atteindre désormais une moyenne d'un an, hors conseils des prud'hommes où la situation est encore plus critique puisque l'on frôle les dix-huit mois. Il n'y a pas de confiance possible dans la justice, si on laisse perdurer une telle situation de thrombose. Il y a ensuite la justice pénale. Arrêtons-nous-y un instant, puisque c'est l'objet principal de ce texte. Entre la première instance et l'appel, il faut plus de deux ans pour traiter les affaires de délinquance, soixante mois pour les affaires criminelles. C'est beaucoup trop. La réponse pénale est trop lente, elle n'est pas adaptée aux exigences d'une politique répressive efficace. D'abord, il y a la réalité de la société : la violence ne cesse de s'aggraver- n'est-ce pas, monsieur le garde des sceaux ? ... -, plus encore vis-à-vis des agents en charge de la sécurité de nos concitoyens. Incontestablement, la France doit faire face à une forte augmentation des violences sur les personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, dis, monsieur le garde des sceaux, non, c'est le Président de la République au mois d'avril dernier, vous l'avez lu comme moi. Croyez bien que ce constat d'échec après quatre années de mandat me navre tout autant que lui et qu'il désole plus encore nos concitoyens exposés à cette aggravation de la violence. Je ne crois pas qu'on les rassurera en filmant le déroulement des procès ou en remplaçant le rappel à la loi par l'avertissement pénal probatoire. Ensuite, cette insécurité aurait normalement dû donner lieu à une amélioration de notre système pénitentiaire. Force est de constater, malheureusement, en ce qui concerne les constructions de prisons, que les engagements n'ont pas été tenus. Monsieur le garde des sceaux, vous vous dites « ulcéré » du procès qui est fait au Gouvernement à propos des 15 000 places de prison que le Président de la République s'est engagé à construire pendant son quinquennat.

de travaux engagés par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux du précédent quinquennat ; 650 places sont en cours de réalisation.

cette carence dans le respect des engagements qui sont au coeur d'un mandat présidentiel posent un véritable problème démocratique. Enfin, il y a la question du budget. L'augmentation des moyens de la justice est réelle, est réelle, il faut le reconnaître, mais elle aura été insuffisante au départ- cela ne sera pas rattrapé -, irrégulière sur la durée, avec une sous-consommation de crédits qui constitue une anomalie grave dans le fonctionnement de l'État. et de réforme pour la justice a été votée tardivement. Elle prévoyait une augmentation de crédit de 23 % en cinq ans. Nous avons jugé que c'était insuffisant, qu'il fallait atteindre si possible 30 %, nous ne l'avons donc pas votée. Vous avez décidé de rétablir la trajectoire que nous souhaitions, nous ne pouvons pas vous le reprocher, nous en sommes heureux. Pour autant, nous ne pouvons pas vous laisser dire que l'effort fait pour la justice permet une remise à niveau, telle qu'elle serait nécessaire pour le bon fonctionnement de la justice. Je l'affirme ! En effet, on ne rattrapera pas les sous-dotations des premières années du quinquennat- cet argent qui n'a pas été dépensé ne le sera plus.

fait que la bataille budgétaire sera entièrement à recommencer au second semestre 2022. Il sera alors trop tard pour tenir la trajectoire budgétaire de 2022. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter de voir les crédits votés, il faut regarder quel aura été

au service d'une rénovation en profondeur de la justice. Nous sommes très nombreux ici à penser que la justice doit cesser d'être un enjeu de débat politique. Nous sommes prêts à contribuer, comme en matière de politique étrangère ou de défense nationale, à ce que des consensus se forgent pour que cette grande fonction régalienne soit mise à l'abri des surenchères et cesse d'être le domaine des bateleurs d'estrade. C'est dans cet esprit que nos rapporteurs ont travaillé, pour essayer d'améliorer votre texte. C'est aussi dans cet esprit que mon groupe soutiendra les efforts de la commission des lois. Même avec ces améliorations, ce n'est certes pas le texte que nous aurions fait si nous avions pu le faire seuls, mes chers collègues. J'ai en particulier les plus grandes réserves sur le fait de filmer des audiences, parce que je suis sensible à l'émotion des victimes comme à la vulnérabilité des accusés, qui sont présumés innocents, et je crains fort que cela n'amène des biais dans la sincérité et l'authenticité des débats judiciaires, et que certains n'en viennent à se servir du tribunal comme d'une tribune. Cependant, le Sénat n'est pas une chambre d'obstruction, monsieur le garde des sceaux, mais de construction. Il sait qu'il ne peut à lui seul faire la loi, et il a donc toujours à coeur d'aborder la discussion des textes avec le sens du compromis, qui permet de trouver des accords consolidant les points qui lui paraissent essentiels- nous vous les signalerons et nous sommes certains que vous contribuerez à une bonne entente avec l'Assemblée nationale. La parole

Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire » : voilà un titre qui sonne comme un aveu ! Mais vous l'avez dit vous-même, monsieur le garde des sceaux, et le sondage commandé par la commission des lois le prouve : les Français n'ont plus confiance dans leur justice. une situation regrettable pour une institution qui est pourtant au coeur de notre pacte social. Les causes de ce désamour sont multiples délais trop longs ; méconnaissance du fonctionnement judiciaire et de ses acteurs ; incompréhension par le grand public de la sévérité, ou du manque de sévérité, des peines prononcées questionnement sur l'exécution de ces peines ; gestion, prévention de la récidive ... La liste est longue, malheureusement. Oui, donc, sur le principe, ce texte est bienvenu. Atteint-il son objectif ? Dans un premier temps, il entend redonner confiance en montrant la justice en action à travers l'enregistrement et la diffusion d'audiences. De prime abord, l'idée m'a paru bonne.

Quel impact auront donc les caméras sur le comportement et la parole des victimes, des témoins, des accusés, mais aussi des procureurs, des juges ou des avocats ?

Vous vous adressiez donc à ces personnes autant qu'à moi. Qu'en sera-t-il dans une session d'assises ? Non, tout ne peut pas être tout le temps filmé, et nos deux rapporteurs, dont je salue ici le travail de grande qualité, ont défini ce qui relève d'un intérêt public, dont l'enregistrement est utile, et affirmé le principe de gratuité, pour éviter toute recherche de surenchère. Rien de tel, à mon sens, qu'une bonne série télévisée, bien documentée, pour faire connaître le métier.

avec l'article 2, qui vise à limiter la durée de l'enquête préliminaire à deux ans, prolongeables d'un an sur décision du procureur. Ce délai semblerait déjà respecté pour 92,7 % des enquêtes préliminaires. Seules 3,2 % d'entre elles dureraient au-delà de trois années. Je dois avouer que ces chiffres me surprennent vraiment, et je crains que la plupart des clôtures ne soient des déclarations sans suite, faute de pouvoir engager les suites en question. Heureusement, l'article exclut de son champ d'application les enquêtes antiterroristes et le crime organisé. Mais il est également un domaine où une enquête prend toujours du temps, les enquêtes financières, ne serait-ce que parce qu'il y a quasiment systématiquement un compte étranger dans l'affaire, mais aussi à cause du manque d'officiers de police judiciaire spécialisés dans la matière. L'extension du délai préconisée par nos rapporteurs en matière de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment est donc la bienvenue. Autre sujet qui a fait causer ou qui fait lire : la suppression du rappel à la loi introduite par nos collègues de l'Assemblée nationale. Il a suffi de le supprimer pour en découvrir toute l'utilité toute l'utilité ! En lisant hier, j'ai pris connaissance de la mesure que vous souhaitiez nous soumettre, l'avertissement pénal probatoire. Le journaliste ne semblait pas avoir compris qu'il fallait encore que nous la votions ... Mais vous avez raison d'avoir eu confiance et d'employer le futur plutôt que le conditionnel, car cette proposition mérite que l'on vous suive.

Mais pendant que les juges seront en train de siéger dans des cours criminelles que l'on généraliserait, ils ne seront ni aux assises ni dans leur bureau. Comment développer des cours criminelles sans se poser la question des moyens à leur consacrer ? Certes, les moyens ont été augmentés

Passons à la pénitentiaire : que du bon ! La fin des remises de peine automatiques était souhaitée par nos concitoyens, et j'ai pu me rendre compte qu'elle était également bienvenue pour les magistrats et les personnels pénitentiaires. Tout le monde serait d'accord, semble d'accord, alors allons-y Un point de vigilance, toutefois, sur les courtes peines qui pourraient partir de la mesure. Autre bonne mesure, le contrat d'emploi pénitentiaire. La peine, c'est la prison, pas le travail sans règles claires. Celles-ci sont mieux définies, on sait qui juge en cas de conflit : c'est un véritable progrès. Enfin, le titre V porte sur le renforcement de la confiance du public dans l'action des professionnels du droit, car la justice, ce ne sont pas que les tribunaux et les juges. Ce sont aussi les notaires, les avocats ou les nouveaux commissaires de justice, regroupant les métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Créer des codes de déontologie devrait permettre de rassurer les justiciables en montrant qu'il n'y a pas les intouchables, d'un côté, et les petits à la merci d'une justice partiale, de l'autre. Souvent, on a pu entendre que les notaires protégeaient les notaires ou les huissiers, les huissiers, par exemple. C'est pourquoi la création d'une phase préalable de conciliation pour les réclamations des usagers, ainsi que la possibilité pour ces derniers de saisir directement la juridiction disciplinaire, ce qui est impossible aujourd'hui, sont des signes positifs et des avancées nécessaires. En définitive, il en faudra probablement plus pour rétablir un véritable lien de confiance entre les Français et leur justice. Pour autant, les avancées que ce texte comporte sont les bienvenues. Elles ont été qui plus est enrichies par nos rapporteurs. Le groupe centriste votera donc ce projet de loi.

il y avait 8 427 magistrats au 1 janvier 2017. Nous en sommes à 9 090 C'est vrai, et c'est incontestable, et 52 magistrats supplémentaires viendront abonder ce nombre. De plus, naturellement, nous pourvoirons aux départs à la retraite.

Je demande à M. le garde des Sceaux et à nos collègues sénateurs de bien vouloir baisser d'un ton dans la forme et sur le fond. Bien sûr, madame la présidente.

mais il est faux de dire que les stocks ont augmenté parce que nous ne les aurions pas traités. Ils ont augmenté parce qu'il y a eu ce qu'on ne peut pas encore oublier, même si on peut s'exprimer maintenant sans masque à la tribune : la covid-19, à laquelle s'est ajoutée une grève des avocats qui a duré six mois.

J'étais encore hier à Nanterre, où la présidente du tribunal judiciaire m'a dit à quel point les stocks diminuaient. Pourquoi ? Parce que nous avons envoyé en masse des personnels, pour le civil comme pour le pénal. Pour le civil, ce sont des juristes assistants. Quand un juriste assistant est aux côtés d'un magistrat, deux fois plus de décisions sont rendues dans le même temps. J'en viens aux établissements pénitentiaires. En fait, vous avez fait le tour

Lutterbach, tout neuf, et si vous allez, monsieur le sénateur Bas, à Caen, en Avignon, à Meaux, à Lille, à Osny, et j'en oublie, vous verrez les 7 000 places qui seront livrées en 2022-2023. Il faudra

et tant que vous ne reconnaîtrez pas que nous en avons fait plus pendant cette mandature que vous durant de bien plus nombreuses années. Je termine, mais souffrez que je vous réponde ! Vous voudriez que je vienne à Canossa, la tête baissée, pour dire que nous n'avons rien fait ? Mais c'est une plaisanterie ! Souffrez que je vous réponde ! Nous souffrons ! Vous me faites le reproche, monsieur le sénateur Bas, de ne pas avoir traité la justice civile dans mon projet de loi. C'est faux, et je vais vous dire pourquoi. Nous Nous traitons d'abord de la simplification de la procédure pour rendre exécutoire un acte d'avocat dans le cadre d'une médiation. Vous savez à quel point c'est important pour les justiciables, parce que cela permet d'aller vite, et que les justiciables, comme ils ont participé à la décision de justice qui les concerne,

calmement, tranquillement, avec- c'est l'objet d'un des amendements que j'aurai l'honneur de présenter -un débat obligatoire après la projection avec des professionnels, au cours duquel on expliquera ce qu'est un témoin, un témoin, un avocat général, une expertise ADN, un conseil de prud'hommes ... Quand on a connaissance des choses, on peut appréhender la réalité qu'on ne connaît pas forcément. Vous, vous connaissez la justice, vous connaissez la règle de droit. Moi aussi,

La médiation, aussi, est de nature à rétablir un peu la confiance. Bien sûr qu'il reste des choses à faire. Mais quel est le garde des sceaux qui serait suffisamment imbécile et arrogant pour prétendre qu'il a tout réglé ? Ce ne sont que de petites briques, mais ce n'est pas rien d'avoir confiance dans son avocat, de savoir qu'on ne va pas violer le secret qui vous unit à lui quand vous êtes un justiciable. Ne pensez-vous pas que c'est de nature à rétablir la confiance, quand on sait que le secret a été complètement balayé ? Le président Hollande avait promis au bâtonnier de Paris, à l'époque, de rétablir le secret : il n'a jamais rien fait

correctement et que, si vous lui reprochez de ne pas l'avoir fait, le différend sera jugé par des juges impartiaux ? C'est pour cela que j'ai demandé l'échevinage, avec la présence d'un magistrat professionnel. Les notaires ont appelé cette réforme de leurs voeux- les avocats aussi d'ailleurs, pour dire vrai, et les huissiers de justice Voilà donc de petites choses, monsieur le sénateur, qui peuvent vous sembler infimes, mais qui me semblent importantes pour rétablir la confiance. Pas toute la confiance, c'est vrai,

de l'écriture, du calcul, pour les plus modestes, pour les plus petits d'entre nous. Quand je l'ai préparé, j'ai rencontré une éducatrice qui m'a dit que, pour certains gamins, se lever le matin est un effort. Cet effort devra être pris en considération

Mais ce que j'ai dit, lorsque j'étais avocat, c'est que je ne voulais pas de cette cour départementale, parce que je pensais qu'elle allait balayer la cour d'assises traditionnelle, à laquelle j'étais extrêmement attaché. Et puis, je suis devenu ministre, et que m'a-t-on dit ? Premièrement, que les magistrats étaient satisfaits de cette nouvelle juridiction. Deuxièmement, que les avocats étaient satisfaits de cette juridiction- à l'exception de quelques braillards qui se sont immédiatement levés pour dire que je reniais mon ancienne robe d'avocat. Troisièmement, que le taux d'appel était de dix points inférieur au taux d'appel que l'on constatait dans le cadre des cours d'assises traditionnelles. Quatrièmement, que cela permettait une fois pour toutes de régler la correctionnalisation des viols, que les victimes ne voulaient plus voir. Cinquièmement, que les audiencements étaient beaucoup plus rapides.

j'ai décidé de la maintenir. Vous m'en faites également le reproche ! Je dois ajouter que, contrairement à ce que vous avez dit, la souveraineté populaire, je l'ai renforcée. Dans le système que j'ai connu avant de devenir ministre, en cour d'assises traditionnelle, un homme pouvait être condamné en l'absence d'une majorité de voix du jury populaire pour le condamner. C'était une première historique dans notre pays et la cour d'assises n'était

dont une sera compensée en janvier. Le procureur général dispose de 5 magistrats placés pour faire face aux vacances. Sur les 130 fonctionnaires, 9 postes sont vacants, soit 6 %.

monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire vise à restaurer la confiance des Français dans la justice. Le titre I contient des dispositions relatives à l'enregistrement et à la diffusion des séances. Il autorise notamment, l'article 1, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience pour un motif d'intérêt public en vue de sa diffusion. Néanmoins,

ou reconstitutions. Lors de la discussion de la proposition de loi améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, le 4 février 2021, j'ai proposé deux amendements portant sur la possibilité pour une personne interrogée de se voir délivrer une copie de son procès-verbal signé par les deux parties. Le but serait de pacifier les relations entre personnes entendues et personnes dirigeant l'interrogatoire. Les arrestations et les auditions sont une source de stress, et parfois de conflits, et cela rend d'autant plus difficile le travail de la justice dans sa recherche de vérité et d'authenticité. La justice étant indépendante, il convient de la rendre la plus transparente possible, en permettant aux citoyens entendus de vérifier leurs déclarations. Actuellement, seule l'autorité enquêtrice dispose de ce droit. Par ailleurs, des cas de modification de déclarations ont déjà été relevés dans le cadre de différentes affaires, la plus célèbre étant celle de Jacques Chirac. Notre Constitution garantit l'indépendance de la justice et l'égalité de tous. Ce genre de manquements désavantage la défense des citoyens. Aussi, je souhaiterais qu'en votre qualité de ministre de la justice, représentant le Gouvernement et porteur de ce projet de loi, vous puissiez intervenir sur les articles 114 et 60-1 du code de procédure pénale, afin qu'une copie du procès-verbal signé puisse être remise aux personnes entendues, ou que celles-ci soient autorisées à photographier leurs déclarations. Le grand avocat que vous êtes, monsieur le garde des sceaux, devrait comprendre et apprécier ma démarche en faveur de la défense. La parole Madame la présidente, permettez-moi d'émettre une réserve sur l'article 1 du projet de loi. Si je comprends l'ambition pédagogique de faire connaître aux Françaises et aux Français le fonctionnement de la justice, je me demande en revanche jusqu'où peut aller cette captation. Il ne faudrait pas transformer les prétoires en justice spectacle.

Les parties, avant de donner leur accord, doivent être éclairées scrupuleusement sur le déroulement et les motifs de l'enregistrement. Ainsi, je demande que l'on précise davantage le motif d'intérêt général, qui me semble bien trop vague. Concilier le respect des droits individuels des acteurs d'un procès et le droit à l'information du public a toujours été en débat. Il est donc nécessaire d'inviter le législateur à se montrer plus précis sur l'objectif visé visé pour déterminer ce qui pourrait relever de l'intérêt public. Nous devons justifier précisément en quoi l'enregistrement sonore audiovisuel des audiences mériterait d'être autorisé,

personnelles, au respect du droit à l'image et à la vie privée, autant de questions qui méritent débat ? Ce projet de loi ne doit laisser place à aucune ambiguïté, puisqu'il s'agit de renforcer la confiance des Français dans notre justice. Nous devons être à la hauteur de cette mission.

à la télévision ou sur internet. L'intention est certes louable : faire entrer la justice dans le salon des Français. Mais la médiatisation aura bien d'autres conséquences ... Trois en particulier me viennent à l'esprit. D'abord, un enregistrement diffusé peut faire l'objet de toutes sortes de montages ou de manipulations. Les exemples ne manquent pas sur internet. Ensuite, tout le monde n'a pas l'habitude des caméras, On peut imaginer que certains participants au procès manquent de spontanéité, ce qui va inévitablement nuire à la liberté des débats. lors de la discussion générale que vous ne souhaitiez pas faire de justice spectacle, mais force est de constater que la télévision laisse de plus en plus de place au spectacle. J'ajoute que la transparence existe déjà, puisque tout citoyen peut aujourd'hui assister à une audience. C'est parce que cette future médiatisation des procès fait débat, autant dans notre assemblée que dans le monde juridique, que je demande une expérimentation pour une durée de cinq ans. Nous regrettons comme d'autres la précipitation avec laquelle est présenté ce projet visant à libéraliser l'enregistrement et la diffusion des audiences sans une analyse approfondie de l'expérience acquise, notamment dans les autres pays européens qui l'autorisent déjà.

C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la mise en oeuvre d'une période d'expérimentation préalable concernant l'enregistrement et la diffusion des audiences, ainsi que la remise par le Gouvernement d'une évaluation complète du dispositif avant toute généralisation. Au regard des enjeux et de la complexité du sujet, qui a tout de même fait l'objet de plusieurs groupes de travail et de réflexion par le passé,

proposé dans ce projet de loi est un vrai bouleversement institutionnel, dont les effets ne sauraient naturellement être prédits. Comment réagiront nos concitoyens, les juridictions, les prévenus, les parties civiles ? Chacun le sait dans cet hémicycle : être filmé n'a rien de neutre, et personne ne peut croire qu'en matière de justice, comme ailleurs, le film d'un procès pourrait correspondre à une transcription objective. Il en résultera une transcription télévisuelle montée en fonction des besoins, d'autant que, comme l'indique le texte, la diffusion pourra être intégrale ou partielle. Bref, tout cela ne doit pas être confondu avec la publicité habituelle de notre justice, que le Conseil d'État a très tôt érigée en principe général du droit, tout en lui fixant comme limite le risque de désordre de nature à troubler la sérénité de la justice. Or, de ce point de vue, nous ne savons pas les effets que pourront produire les diffusions. Nous devrions donc nous engager sur une voie plus prudente, ce que permet cet amendement, qui vise à rendre le dispositif expérimental. Quel est l'avis de la commission ? Cet article 1 sur l'enregistrement et la diffusion des audiences crée une nouvelle exception à l'article 38 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, autorisant donc l'enregistrement et la diffusion pour un motif d'intérêt public.

ouvrir la justice aux Français et à leur faire mieux connaître son fonctionnement, offre un certain nombre de garanties, que nous avons par ailleurs renforcées. Il ne prévoit la diffusion que dans des délais allongés, notamment une fois que l'affaire est que toutes les voies de recours sont épuisées, ce qui peut prendre un certain temps. Mettre en place une expérimentation limitée à cinq ans ne permettra pas forcément d'évaluer toutes les

du décret. Au demeurant, ce n'est pas une idée nouvelle. Robert Badinter y avait déjà songé. Un certain nombre de procès avaient déjà été filmés,

En ayant accès à ces derniers, nos concitoyens justiciables pourraient avoir une idée un peu moins confuse et un plus précise de leurs droits et du déroulement d'un procès, à condition bien évidemment que le procès soit sélectionné avec le plus grand soin, qu'il s'agisse d'affaires du quotidien, et non de grandes affaires fortement médiatisées.

: La parole est à M. Hussein Bourgi. Au regard des objectifs d'éducation civique prêtés à l'enregistrement et à la diffusion des audiences à la télévision, nous proposons que les éventuelles diffusions aient lieu exclusivement sur les chaînes de télévision du service public. en effet que celles-ci sont plus à même de remplir cette mission pédagogique, d'autant qu'elles sont moins soumises aux pressions liées à la course à l'audimat. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement

La décision finale et souveraine appartient au président du tribunal des conflits, au vice-président du Conseil d'État, au Premier président de la Cour de cassation ou au Premier président de la Cour des comptes. Quel

Il vise, d'une part, à aligner le régime d'autorisation prévu pour les juridictions judiciaires et administratives de premier ressort et d'appel sur celui prévu pour les cours suprêmes, en prévoyant un avis simple, et non une proposition du ministre de la justice. Il vise par ailleurs à procéder à une amélioration rédactionnelle relative à l'autorité décisionnaire, afin de bien viser l'ensemble des audiences.

et non uniquement aux parties au litige, comme le prévoit le texte actuel. Il s'agit là notamment d'une préconisation de l'Union syndicale des magistrats (USM) et du Syndicat de la magistrature, qui vise à garantir que le droit à l'image soit respecté pour chacun, y compris pour les professionnels présents à l'audience. La mission des professionnels qui rendent la justice ou concourent à son exercice ne comporte en effet aucune obligation de passer à la télévision, même floutés, d'autant que les garanties d'anonymat sont très restreintes dans le projet de loi. Il s'agit également de veiller au consentement des personnes présentes lors de l'audience, si celle-ci est filmée. Il aurait d'ailleurs été nécessaire de permettre un droit de rétractation après l'enregistrement de l'audience pour toutes et tous, celui-ci n'étant pour l'heure réservé qu'aux personnes jugées, aux plaignants et aux témoins, et de fixer un délai suffisant d'information, comme le souligne le Syndicat de la magistrature. Une personne est-elle véritablement en mesure d'apprécier les enjeux si la demande lui est soumise le matin même de l'audience ? Quel Quel est l'avis de la commission ? Votre amendement personnes présentes lors des audiences qui ne sont pas publiques. Actuellement, le texte ne prévoit que l'accord des parties. Les autres personnes, qui sont des professionnels de la justice principalement, des témoins ou des experts, sont donc enregistrées sans leur accord, mais peuvent s'opposer à la diffusion de leur image et demander l'anonymisation de leur participation. Le dispositif nous paraît équilibré. Imposer un accord à tout le monde rendrait

vise à permettre au ministère public, lorsqu'il est représenté, de s'opposer à l'enregistrement dès lors qu'il considère que sa diffusion pourrait porter atteinte aux intérêts des parties. Il pourrait aussi s'opposer, dans un délai de quinze jours et à l'issue de l'audience, à sa diffusion.

de loi énonce que « les modalités de l'enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées

En conséquence, l'enregistrement d'une audience ne doit pas permettre de retranscrire ces échanges ou de les restreindre, par crainte et anticipation des parties d'être entendues.

69 visant à expérimenter ce dispositif d'audiences filmées, nous proposons cet amendement plusieurs aménagements pour améliorer le dispositif. D'abord, nous souhaitons prévoir la diffusion des enregistrements au minimum un an après que l'affaire a été définitivement jugée,

Toute autre solution accroît le risque de verser dans la justice spectacle, qui n'est en rien propice à la sérénité des débats. Par ailleurs, nous estimons que le meilleur canal de diffusion serait une page spéciale du le site internet

prévoit des diffusions à l'image de la diversité des audiences. En effet, ces diffusions ne sauraient être focalisées sur le seul procès pénal, qui peut être instrumentalisé à des fins politiciennes.

ainsi que les conditions souvent indigentes dans lesquelles les professionnels de la justice sont amenés à travailler. Quel est l'avis de la commission ? La commission

fondamentaux de notre société. L'alinéa 11 prévoit en l'état que « la diffusion est réalisée dans les conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d'innocence. » Nous proposons, par cet amendement, d'y ajouter le respect de l'anonymat, d'autant que la garantie explicite d'un tel principe peut également servir à assurer la sécurité de toutes les personnes participant au procès. En effet, nous pouvons facilement imaginer qu'une personne puisse, par

parole est à M. Jean-Yves Roux. Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 prévoit un certain nombre de garanties pour les acteurs de l'audience. Je pense par exemple au fait que l'image et les autres éléments d'identification des personnes enregistrées

Le Gouvernement avait initialement précisé que les audiences pouvaient être filmées pour un « motif d'intérêt public